Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des

Il y a la manière brutale et la dissimulation, et il y a le montant- 52 milliards d'euros, ce n'est pas rien ! Mais l'essentiel n'est pas là. Il est dans l'attitude des États-Unis, qui ont contraint l'Australie, comme ils avaient obligé les Suisses à acheter leurs chasseurs F-35 plutôt que le Rafale. Biden, que nous avions porté aux nues, fait au fond ce que fait tout président des États-Unis. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les États-Unis montrent le peu de cas qu'ils font de leurs alliés, ou prétendus tels : rappelez-vous Obama et la Syrie en 2013 En l'occurrence, on peut se demander si les États-Unis ne se sont pas tiré une balle dans le pied. Ils perdent la confiance des grands pays européens, qui nous ont manifesté leur soutien hier à l'occasion de

nous aurions pu participer à une stratégie globale pour la région, mais y a-t-il encore une alliance devant tant de duplicité ? Madame la ministre, mes questions sont les suivantes. Quelle stratégie alternative peut-il y avoir pour la France, qui cherche à construire une alliance régionale

? Enfin, notre coopération militaire avec la Grande-Bretagne- je pense aux accords de Lancaster House -peut-elle survivre à ce Trafalgar ?

de saluer votre engagement sans faille, au cours de ces dix-sept dernières années, sur les questions internationales, européennes et de défense. Vous le savez, la France

espace maritime. Nous ne sommes pas seuls, monsieur le sénateur, dans la zone indo-pacifique. Nous y avons des partenaires importants : l'Inde, le Japon, la Malaisie ou encore l'Indonésie.

Cette stratégie trouvera un écho dans la « Boussole stratégique », ce premier livre blanc de la défense européenne qui sera l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne, qui

où ses intérêts sont en jeu. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Français et pour les Européens. La

Bien sûr, nous condamnons, comme vous, les agissements de nos alliés américains, britanniques et australiens, mais force est de constater que cette affaire dite des sous-marins australiens en dit long sur votre gouvernance et votre bilan.

au premier rang desquels les États-Unis ? C'est en effet une question sérieuse qui me paraît nécessiter la mobilisation de chacun Les Français auront l'occasion de s'exprimer sur les débats de politique intérieure dans quelques mois. Alors, si vous le voulez bien, revenons à l'affaire qui nous intéresse

La parole est à M. Éric Gold, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. chargée des sports. Madame la ministre, la pratique sportive a été considérablement affaiblie depuis le début de la crise sanitaire. Les clubs sportifs amateurs sont à la peine : la chute du nombre de licenciés et de bénévoles met en péril leurs finances et l'organisation des compétitions. La baisse de l'activité physique a été qualifiée de bombe à retardement sanitaire dans un rapport de l'Assemblée nationale. Si la réponse du Gouvernement, par l'intermédiaire du Pass'Sport, apparaît comme une initiative intéressante, avec une aide de 50 euros sur l'adhésion à une association sportive pour les 6-17 ans sous certaines conditions, l'enveloppe dédiée de 100 millions d'euros semble largement insuffisante pour toucher les plus de 5 millions de jeunes concernés. En outre, les débuts du Pass'Sport sont particulièrement timides- Si certains attendent de savoir, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, si les compétions auront bien lieu cette année, d'autres se heurtent aux difficultés des associations dans la mise en place de la mesure. L'Agence nationale du sport demande en effet aux clubs la création d'un « compte asso » pour le remboursement des 50 euros qui ne sont pas demandés aux bénéficiaires du Pass'Sport.

outre, dans un pays où 17 % de la population est touchée par l'illectronisme, imposer la création d'un compte internet rend nécessairement la mesure moins populaire. Le décret, publié le 10 septembre, en est à ses tout débuts, mais c'est maintenant que se joue la saison, c'est maintenant que se constituent les équipes et que les associations ont enfin l'occasion de sortir la tête de l'eau. Je présenterai, le 14 octobre, avec mes collègues du groupe du RDSE, une proposition de loi visant à créer une aide supplémentaire sur les adhésions sur les adhésions aux associations sportives, culturelles et récréatives, et à relever la réduction d'impôt en vigueur sur les dons à ces associations. Aussi, madame la ministre, quelles mesures complémentaires et quelles aides aux associations le Gouvernement compte-t-il mettre en place pour soutenir les bénévoles et le sport amateur en général ? La parole

sur l'adhésion sportive pour un jeune sur deux incite fortement les enfants et les jeunes à s'inscrire en club, c'est-à-dire à une activité encadrée et sécurisée, essentielle, vous l'avez dit, pour la santé et le bien-être de nos jeunes : 5,4 millions de jeunes de 6 à 17 ans sont concernés et nous recevons les inscriptions de 15 000 enfants directement en ligne.

secrétaire d'État chargée de la biodiversité, il y a quelques jours, au sommet mondial de la biodiversité à Marseille, le Président de la République déclarait dans un beau discours sa détermination à porter haut et fort les enjeux de la biodiversité. Et voilà que nous apprenons que le Gouvernement s'apprête à réautoriser des pratiques de chasse récemment interdites, avec le piégeage traditionnel de plus de 100 000 oiseaux sauvages appartenant à des espèces en déclin, déclin, alors même que le Conseil d'État et la Cour de justice de l'Union européenne ont récemment déclaré ces pratiques illégales et que la France a perdu- rappelons-le -près du tiers de ses oiseaux depuis le début du XXI siècle. Vous n'en serez pas surprise, madame la secrétaire d'État, mais il nous paraît totalement inimaginable de tolérer demain, à nouveau, ces chasses non sélectives. L'Espagne a déjà été condamnée par l'Union européenne sur ce fondement. Certains prétendent que, défendre la chasse, c'est défendre la ruralité,

La majorité des ruraux sont d'ailleurs opposés à ces pratiques de chasse. Les chiffres sont têtus : seuls 26 % des ruraux sont favorables à la chasse telle qu'elle est pratiquée et 70 % des chasseurs sont des urbains- Oui, nous appelons au respect de la ruralité ! Une ruralité bienveillante, vivante et respectueuse de toutes et de tous. Respecter la ruralité, c'est d'abord cesser de soutenir un modèle libéral qui métropolise la France, en détruisant les emplois ruraux. C'est cesser cette agriculture intensive qui met à mal trop de paysans et de paysages. C'est arrêter de détruire les services publics. C'est aussi pouvoir, le dimanche, se promener tranquillement, en paix, en forêt ou sur des chemins ruraux.

débat. Il est évident que personne ne souhaite voir s'installer une agressivité et une tension entre un monde présumé urbain et un monde rural, mondes qui seraient soi-disant incapables de se comprendre et de s'entendre.

La profession souffrait déjà avant la crise d'un manque d'attractivité et de mauvaises conditions de travail. En 2018, on dénombrait un infirmier pour 1 300 élèves. Désormais, avec un infirmier pour 1 800 élèves en Seine-Saint-Denis, il est impossible de travailler correctement. travail des infirmiers scolaires s'est considérablement accrue avec la mise en place des mesures sanitaires et l'augmentation importante des besoins d'accompagnement des élèves affectés par la crise. Autre facteur aggravant, leur rémunération est largement inférieure à celle proposée par les établissements de santé. La situation est telle que 66 % des infirmiers scolaires envisagent de changer de métier et nous savons que nombre d'entre eux ont déjà franchi le pas, accentuant la charge de ceux qui restent, faute de remplaçants. Monsieur le ministre, la situation n'est plus tenable. Vous connaissez le rôle fondamental des infirmiers de l'éducation nationale. Outre leur rôle de soignant, ils sont le dernier rempart contre le décrochage scolaire, la dépression, la maltraitance familiale ou le harcèlement. Leurs missions de prévention de ces risques, d'écoute, de détection des situations d'urgence et d'accompagnement sont indispensables au bon fonctionnement de l'enseignement. Nous ne pouvons faire l'économie d'une juste revalorisation de la profession, au-delà de celle annoncée dans le cadre du Grenelle de l'éducation, qui va dans le bon sens. Cela passe, bien entendu, par une hausse des salaires, mais aussi par une formation adaptée et éventuellement une territorialisation du recrutement dans le cadre d'une réorganisation globale de la santé scolaire. L'égalité d'accès à la santé des élèves est une composante essentielle de l'égalité des chances. Pourriez-vous préciser, monsieur le ministre, les actions que le Gouvernement entend mettre en place pour lutter contre la pénurie d'infirmiers de l'éducation nationale ?

je vous remercie pour cette question, qui permet de mettre l'accent sur les infirmiers et les infirmières scolaires, lesquels, comme vous l'avez très bien dit, représentent un corps essentiel pour l'éducation nationale. Leur rôle est extrêmement

en faveur de l'électronucléaire, en considérant, comme nous l'estimons très largement au sein du groupe auquel j'appartiens, que le nucléaire n'est pas simplement un complément, mais qu'il est surtout une condition de la décarbonation de l'énergie en Europe. Europe. Madame la ministre, vous avez en charge l'industrie. C'est formidable, parce que le nucléaire est, pour notre industrie, un atout fantastique. Oh là là ! La France va présider l'Union européenne pendant six mois et ma question est question est simple : allez-vous convaincre nos partenaires que, dans une situation d'extrême urgence où la transition énergétique est un devoir absolu, il faut nous fixer une priorité qui est de décarboner,

Et lorsque le commissaire Johannes Hahn explique très clairement que les obligations vertes ne seront pas ouvertes- c'est le cas de le dire -au nucléaire, mais qu'il est envisageable qu'elles

Aussi, dans ce moment d'urgence climatique, nous aurions tort de ne pas nous appuyer dessus. C'est clairement la stratégie que nous suivons. Vous l'avez d'ailleurs mentionné, Bruno Le Maire a été particulièrement clair, tout comme le Président de la République ou

de réponse au défi climatique. Cela avait été une négociation portée fortement par le Président de la République. Nous allons continuer avec la taxonomie. Sur ce sujet, nous avons le soutien du commissaire Breton, qui a une vision industrielle pour l'Europe, fondée sur des faits et non sur de la démagogie ou des rêves.

donnée à la neutralité technologique, à une vision industrielle, qui englobe tous les effets pour l'emploi et pour la décarbonation, ainsi qu'à une accélération de cette dernière, parce que c'est l'urgence du moment pour sauver notre industrie, nos emplois et notre climat. La parole est

Les prix du gaz, de l'électricité et du pétrole ne cessent de battre des records. Le gaz s'est renchéri de 300 % et l'électricité de 97 % depuis le début de l'année. En une semaine, l'essence a augmenté de 15 %. Or cette flambée promet d'être durable. Les prix du gaz et de l'électricité sont au sommet, alors que la saison froide n'a pas commencé. Sont en cause la faiblesse des stocks européens et la hausse du prix du CO2.

elles ont déjà commencé à en souffrir -, ensuite pour les ménages, dont la facture énergétique devrait bondir de 10 % au début de l'année prochaine, et, enfin, pour l'ensemble de l'économie, car cette flambée pourrait être responsable d'un demi-point d'inflation dans la zone euro en fin d'année. le ministre, le chèque énergie, réactivé par le Gouvernement, n'est pas à la hauteur du problème. Quelle est la stratégie énergétique de la France ?

comme l'Espagne, où de nombreux tarifs sont indexés sur les cotations journalières et, donc, très exposés à la hausse des marchés, les ménages français sont, par construction, plus protégés face à cette volatilité des marchés. En effet, dans les coûts d'approvisionnement sont pris en compte les tarifs réglementés de vente, qui comprennent une part versée à l'Arenh, ce dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dont le prix est fixe. Les consommateurs bénéficient donc de la compétitivité et de la stabilité des coûts du nucléaire. Ensuite, les tarifs réglementés comprennent aussi une part d'approvisionnement aux marchés en partie lissée sur vingt-quatre mois, ce qui est un autre facteur de stabilité.

permettrait, certes, d'augmenter sa pondération dans le calcul des tarifs réglementés en 2022 ; mais une décision unilatérale présenterait également des risques juridiques trop importants à court terme et qui pourraient rendre cette décision inopérante. Le Gouvernement considère donc que cette solution n'est

Les États-Unis ont choisi de faire de la zone indo-pacifique un espace de confrontation directe, y compris sur le terrain militaire, avec la Chine, et ils ne toléreront leurs alliés que sous leur commandement et à leur seul profit. profit. Ils sont prêts pour cela à encourager une escalade dans le surarmement de la région, quitte à disséminer des technologies militaires nucléaires utilisant de l'uranium enrichi, et ce au mépris des engagements de non-prolifération. Enfin, ils envoient par la même occasion à leurs alliés de l'OTAN un message d'alignement brutal, qui vise directement quiconque en Europe envisagerait de s'écarter du rang. Madame la ministre, est-ce l'intérêt de la France et de l'Europe de continuer à s'aligner derrière de tels projets ? Est-ce l'intérêt de la France de continuer à participer au commandement militaire intégré de l'OTAN, dont les États-Unis viennent de nous dire qu'ils veulent être les seuls patrons ? Est-ce l'intérêt de la France de tourner toute son industrie militaire vers la course à l'exportation d'armes, en quémandant notre « part du gâteau » auprès des Américains ? Est-ce l'intérêt de la France et des Européens de courir dans ces conditions après une Europe de la défense définie comme un pilier européen de l'OTAN, un pilier auquel on dénierait toute autonomie stratégique maîtrisée par les Européens eux-mêmes ?

Je pense évidemment à l'aventurisme turc en Méditerranée ou bien au retrait précipité et non concerté d'Afghanistan, dont nous avons vu les dramatiques conséquences. L'attitude des États-Unis à l'égard du programme des sous-marins, évoquée voilà quelques minutes, est une nouvelle illustration du constat que nous faisons depuis des mois mois : aujourd'hui, le dialogue politique est inexistant au sein de l'Alliance atlantique. Alors, quelles conséquences faut-il en tirer ?

en témoignant de sa solidarité auprès des États baltes dans le cadre d'opérations de présence de l'OTAN. Toutefois, la raison d'être de l'OTAN, non pas la confrontation avec la Chine, mais la sécurité transatlantique, et c'est ce que nous devons rappeler aux États-Unis. C'est donc dans cette logique que les alliés ont décidé, sur notre initiative, ainsi que sur celle de l'Allemagne, d'engager une révision du concept stratégique de l'Alliance. Ce travail nous permettra de clarifier celui-ci, et c'est nécessaire, dans la perspective du prochain sommet de Madrid, et, surtout, de le faire en cohérence avec la « Boussole stratégique », ce travail lancé par les Européens pour renforcer l'Europe de la défense. Pour terminer, monsieur le sénateur, je dirai qu'être allié ce n'est pas être l'otage des intérêts de l'autre.

du Gouvernement lors des différents référendums sur le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans le périmètre de la République ait contribué à ce résultat, nos alliés ayant sans doute besoin de s'assurer de la pérennité de la présence de

l'État est neutre pour organiser le scrutin ; le gouvernement de la République, lui, peut témoigner d'une orientation ou d'une préférence. Le Président de la République, en tant que chef de l'État, l'a fait lors de son discours à Nouméa, devant le théâtre municipal, et le Premier ministre Jean Castex, ici présent, l'a fait

qu'au fond la Nouvelle-Calédonie n'avait pas d'ennemis, que la zone était calme et qu'une Kanaky indépendante n'aurait pas besoin d'armée. La guerre froide n'a eu que très peu d'impact sur les accords de Matignon-Oudinot en 1988. Le contexte qui a entouré les accords de Nouméa, en 1998, a peu souffert d'ingérences étrangères.

de la parole de la France qui est en jeu. Il s'agira de définir un destin pour la Nouvelle-Calédonie le 13 décembre au matin, en espérant, monsieur le sénateur, que la campagne présidentielle ne vienne pas politiser excessivement un dossier très complexe. C'est en tout cas le voeu que je forme, et je pense que le Sénat aura à coeur

Je suis désolé de vous le dire ainsi, mes amis : c'est facile de donner des leçons de morale en déclarant que l'OTAN est en situation de mort cérébrale, mais c'est un peu plus compliqué

avait raison de demander cette révision de la LPM, qui nous aurait permis d'avoir un débat au fond. Vous êtes en train de réussir cette performance merveilleuse du « en même temps

des collégiens nés en 2010 sont la cible d'une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux menée par des collégiens plus âgés. Ce nouveau phénomène, apparu notamment sur les réseaux TikTok et Twitter, qui encourage les insultes et les menaces envers les enfants nés en 2010, s'est également prolongé dans les cours de récréation, où certains élèves ont été agressés. Le harcèlement, notamment le cyberharcèlement scolaire, qui ne connaît, lui, aucune limite géographique ni temporelle, est un véritable drame pour les enfants qui en sont victimes et peut avoir des conséquences dramatiques. Comme vous le savez, monsieur le ministre, le Sénat a mis en place une mission d'information sur le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement, laquelle doit rendre ses conclusions cette semaine. Nous avons donc rencontré de nombreux acteurs pour mieux comprendre et tenter de mettre un terme à ce phénomène. Il est en effet de notre responsabilité de protéger les élèves d'aujourd'hui, qui seront les citoyens de demain.

Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre concrètement pour éradiquer ce fléau qui touche notre jeunesse, déjà durement éprouvée par les conséquences de l'épidémie de la covid-19 ?

un sujet de société derrière cette question du cyberharcèlement, que je vous remercie de soulever aujourd'hui. La semaine dernière, elle a défrayé la chronique sur des bases totalement absurdes, avec la montée en puissance du hashtag #Anti2010.

Il est essentiel que nous ayons une stratégie d'ensemble sur le cyberharcèlement et c'est ce que nous faisons depuis 2017. En cette rentrée s'applique dans tous les établissements de France le programme Phare, qui est un programme anti-harcèlement, inspiré en partie, d'ailleurs, d'expériences scandinaves, auxquelles vous avez fait référence, et qui conduit à responsabiliser tout le monde, d'abord par la formation

De même, nous responsabilisons les élèves, avec des ambassadeurs contre le harcèlement dans chaque établissement de France. C'est le point le plus important du programme Phare. Une formation spécifique est

j'ai invité l'ensemble des responsables de plateforme à venir me rencontrer lundi prochain, en présence du président du CSA, Roch-Olivier Maistre, qui a des compétences en matière de sanction des acteurs de l'audiovisuel comme des plateformes de réseaux sociaux, de façon à écouter les propositions qu'ils nous font. Nous avons des idées très claires et très précises sur la nécessité d'encadrer beaucoup plus ce qui se passe pour les jeunes sur les plateformes. Nous avons déjà pris des mesures depuis 2017. Je pense à l'interdiction des téléphones portables au collège. Bien entendu, je serai très attentif, dès cette semaine, aux premières conclusions de vos travaux, qui sont évidemment de la plus haute importance. C'est donc la semaine prochaine, après en avoir pris connaissance, que nous franchirons une nouvelle étape dans la lutte contre le cyberharcèlement. La parole

Monsieur le Premier ministre, nous avons réclamé ici, au Sénat, des gestes pour les pieds-noirs, les harkis, les anciens combattants, notamment lors des différentes lois de finances : augmentation des crédits en faveur du monde combattant ; proposition de versements exceptionnels pour les rapatriés. Votre majorité a rejeté systématiquement nos propositions. Soudainement, peut-être- je dis bien peut-être ... -à quelques mois des élections, le souvenir rejaillit opportunément à l'Élysée : le président Macron demande pardon aux harkis au nom de l'État avec une nouvelle loi de réparation. Oui, monsieur le Président de la République, les harkis méritent que leur souffrance soit reconnue. Ils se sont battus pour la France et la France les a abandonnés. Certes, le « en même temps » est votre marque de fabrique, mais ce « en même temps mémoriel » est particulièrement malvenu. Monsieur le Premier ministre, mes questions sont claires. Comment peut-on accuser, comme Emmanuel Macron l'a fait en Algérie, en février 2017, les Français de crimes contre l'humanité et reconnaître en même temps les souffrances de leurs fidèles soutiens ?

Comment s'apprêter à célébrer en grande pompe le soixantième anniversaire des accords d'Évian, alors que cette date marque une défaite pour la France et le début d'un « permis de tuer » ces mêmes harkis que vous prétendez aujourd'hui mettre à l'honneur de l'histoire de France ? pouvez-vous donc prendre l'engagement qu'aucun membre de votre gouvernement ne participera aux cérémonies du 19 mars prochain, pour être enfin cohérent avec vos discours ?

que ces mémoires se parlent, qu'elles soient toutes respectées et qu'elles se respectent entre elles. C'est un objectif ambitieux, et le chemin est difficile, mais je souhaite véritablement, tout comme le Président de la République, que que le soixantième anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie- je sais que vous allez me dire que ce n'est pas la fin ! -soit l'occasion

pour la réplique. Pour nous, chère madame, le devoir de mémoire n'est pas à la carte, au gré des échéances électorales. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire.

Depuis 2016, la sélection se fait en effet à l'entrée en master 1, après l'obtention d'une licence, en cohérence avec le système LMD. Or, parallèlement à l'augmentation considérable des effectifs de licence ces dernières années, l'offre de masters n'a pas été calibrée sur l'évolution de la demande dans les filières où l'obtention d'une licence seule est insuffisante pour accéder au marché du travail. Je pense notamment aux études de droit. Consciente du problème, vous avez annoncé cet été la création de nouvelles places dans les filières en tension. Visiblement en nombre insuffisant, puisque les étudiants sont encore des milliers à se précipiter sur la plateforme gouvernementale « trouvermonmaster.gouv.fr », censée leur obtenir une solution. Or nombreux sont ceux à qui la plateforme ne propose rien de pertinent. Ils sont, de fait, exclus du système. Cette situation vide de son contenu le droit à la poursuite d'études, qui doit pourtant garantir un parcours cohérent. Madame la ministre, que pouvez-vous proposer à ces étudiants ? Plus largement, comment entendez-vous concilier droit à la poursuite d'études et sélection sans les opposer ?

vous le savez, je suis toujours très attentive aux travaux du Parlement en général, de la Haute Assemblée en particulier. Aussi, je me souviens parfaitement que, le 9 septembre dernier, nous avons célébré le cinquième anniversaire de la proposition de loi (PPL) de votre prédécesseur, M. Jean-Léonce Dupont, qui a proposé de manière sèche la sélection à l'entrée du master. Ce texte s'est trouvé prolongé par la loi du 23 décembre 2016, qui a prévu, en même temps que la sélection, le droit à la poursuite d'études. Vous voyez que le « en même temps » a quelques années derrière lui et, probablement, quelques belles années devant lui aussi. Alors, que faisons-nous depuis cinq ans ?

un master, s'ils le souhaitent, à condition qu'on puisse ensuite les insérer professionnellement. Bravo ! La parole

Après sept mois de concertation, de déplacements et d'échanges autour du Beauvau de la sécurité, le mardi 14 septembre dernier, à Roubaix, le Président de la République nous livrait ses propositions pour la sécurité des Français. Il était temps ! Il était temps, monsieur le Premier ministre, quatre ans après l'élection présidentielle, que des mesures soient annoncées ! Entre-temps, de 2016 à 2020, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 36 %. presque 800 agressions par jour ! Les violences à l'encontre des dépositaires de l'autorité publique ont également augmenté de 12 % : il y en a presque 100 par jour Dans notre beau pays, une violence gratuite est commise toutes les 44 secondes ; un refus d'obtempérer, toutes les 30 minutes ! Il était donc temps, monsieur le Premier ministre, à quelques mois des élections, que le Président de la République entende l'appel du Sénat et des forces de sécurité. Simplification des procédures pénales, meilleure prise en charge des victimes, formation et soutien plus performants offerts aux policiers et aux gendarmes : tout cela, nous le proposions déjà en 2018. d'enquête du Sénat sur l'état des forces de sécurité intérieure. La création d'une réserve opérationnelle de la police, c'est aussi une proposition du Sénat, faite en début d'année Vous l'aurez compris, monsieur le Premier ministre : je me réjouis que l'ensemble du travail accompli par notre institution ait été repris. Mais le Président de la République aura du mal à mettre en place ces réformes dans un temps court.

Le Beauvau de la sécurité a été un temps d'échange et de travail direct, sans filtre et continu, qui a permis d'écouter la réalité du terrain et de trouver des solutions concrètes : le ministère de l'intérieur y a apporté un engagement sans faille. À la suite du Beauvau, le Président le Président de la République a entendu les préoccupations des Françaises et des Français, ainsi que celles de nos forces de sécurité intérieure. Il a donc annoncé de nombreuses mesures concrètes, que vous connaissez.

Au-delà de cet engagement budgétaire sans précédent, nous présenterons en début d'année prochaine un projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, texte qui structurera encore davantage notre police, notre gendarmerie

Le continuum de sécurité entre l'État et les maires est fondamental dans notre approche commune de la sécurité des Français. Cela passe par l'augmentation, dès 2021, des moyens dédiés à la vidéoprotection. C'est C'est donc en ce sens, et avec conscience du souci particulier de la Haute Assemblée pour les collectivités locales, que je veux rappeler ici que quatre maires ont participé activement au Beauvau de la sécurité et que l'ensemble des associations d'élus

de répondre aux attentes par rapport à l'évolution des besoins australiens, nous contentant plutôt d'un excès de confiance en nous-mêmes et de propos incantatoires ; cela sera l'objet de la commission d'enquête que nous appelons de nos voeux. Nous ressentons

inquiets pour le devenir de nos industries de défense, qui enregistrent un nouveau camouflet après l'échec de la vente de Rafale à la Suisse. Après un tremblement de terre, outre des ruines, il y a des personnes sous les décombres et des édifices fragilisés. Aussi, madame la ministre, quelles mesures concrètes, économiques et sociales, l'État mettra-t-il en place pour accompagner les salariés, mais aussi ces entreprises qui vont faire face à une rupture de charge brutale et sont plus fragiles économiquement moins armées juridiquement ? Est-il envisageable, notamment, d'avancer les études du programme de sous-marins de troisième génération pour mobiliser les moyens en ingénierie qui vont s'avérer disponibles ?

à Naval Group, ainsi qu'à toutes les entreprises françaises, aux ingénieurs et aux militaires qui, pendant plus de quatre ans, se sont donnés pour ce programme d'armement. Notre industrie navale figure parmi les meilleures du monde. C'est une fierté de cultiver en France des savoir-faire uniques, connus et reconnus, qui permettent à notre marine nationale d'être l'une des meilleures au monde. La rupture de ce contrat, c'est un coup porté à nos emplois. Sans compter les sous-traitants que vous avez évoqués, 650 personnes

s'est traduite par la mise à disposition de logements, de services et d'écoles adaptés aux besoins de ces personnes. ? Eh bien, nous n'allons pas nous laisser faire ! Nous allons aider nos entreprises à passer ce cap, et ce de deux manières. Tout d'abord, en sortant par le haut : les études qui ont déjà été réalisées

aux côtés de Naval Group et des collectivités territoriales concernées pour trouver des solutions et assurer le maintien des compétences. Dans cette perspective, le récent le récent lancement en réalisation du sous-marin nucléaire lanceur d'engins de troisième génération ainsi que les travaux portant sur le porte-avions du futur, grands programmes lancés grâce à la loi de programmation militaire, nous aideront beaucoup.

pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le ministre, la vague épidémique sans précédent de covid-19 qui a frappé les Antilles, dont Saint-Martin, a mis en exergue les fragilités structurelles des systèmes de santé de nos territoires respectifs. Ainsi, si la situation critique qu'a connue notre centre hospitalier Louis-Constant-Fleming est exceptionnelle, elle est néanmoins révélatrice des graves carences dont souffre notre territoire et suscite de légitimes interrogations.

Malgré sa petite taille, c'est le seul recours pour la population de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. À ce titre, il doit être capable de répondre à l'ensemble des besoins en urgence et en première intention pour les soins courants.

De plus, les restrictions horaires de décollage et d'atterrissage des avions- l'un comme l'autre sont impossibles la nuit -peuvent entraîner un important retard de prise en charge et une réelle perte de chance pour nos patients. Oui, on meurt à Saint-Martin faute de disponibilité d'un hélicoptère de la sécurité civile de la Guadeloupe ! Oui, le temps d'attente pour des analyses à l'hôpital est de deux heures au minimum, faute de laboratoire disponible 24

Que comptez-vous faire pour que notre centre hospitalier réponde enfin aux exigences d'un établissement isolé, ce qui garantirait à la population saint-martinoise une prise en charge correspondant aux mêmes standards que ceux qui s'imposent sur le territoire hexagonal en matière d'accès aux soins et d'égalité des chances ?

permettre un meilleur accès aux soins à tous nos concitoyens. Pour maintenir cette promesse républicaine, il est nécessaire de travailler collectivité par collectivité, très finement pour trouver la réponse la plus adaptée.

Nous devons donc tâcher d'apporter la réponse la plus indiquée à ce territoire pour permettre à ses résidents de disposer de l'offre la plus consolidée possible. D'ores et déjà, sur les territoires couverts par l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, nous allons mobiliser 10 millions d'euros pour la première année

que l'on passe en boucle sur les chaînes d'informations : les habitants y perdent parfois des souvenirs, leurs biens, voire un proche ; une fois ces inondations vécues, ils ne se sentent plus jamais en sécurité.

de 21 000 habitants. Alors que les investissements attendus sont considérables, le plafond mobilisable ne sera jamais suffisant pour ces territoires du fait de leurs caractéristiques géographiques et démographiques. La protection de nos concitoyens passe par des investissements lourds, de plusieurs millions d'euros. Pour ne prendre qu'un exemple, la communauté de communes Terre de Camargue est à l'aval de trois bassins versants, qui couvrent près de 20 % du territoire national. Il faut que l'État incarne et finance la solidarité amont-aval dont nous avons besoin. Ma question est donc la suivante : êtes-vous prête à soutenir à une hauteur exceptionnelle le financement des ouvrages nécessaires ? La parole

est suspendue. La séance est reprise. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 23 voix pour, aucune voix contre -à la nomination de M. Serge Lasvignes à la présidence de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

pourrait ainsi être appliquée dans la limite de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. En cas

Alors que la juste rémunération des producteurs agricoles est devenue, à juste titre, une attente de plus en plus forte de nos concitoyens, de nombreux opérateurs fondent leur communication et leur marketing sur cette thématique.

Dans cet esprit, notre amendement vise à mieux lutter contre ces pratiques, sur le modèle du dispositif proposé à l'article 3 par la commission des affaires économiques : en obligeant le Gouvernement à rendre annuellement compte au Parlement de ses actions en la matière dans un rapport public, la mesure proposée vise à faire toute la transparence sur les moyens dont dispose la DGCCRF, sur les mesures prises par le Gouvernement sur ce sujet et à rendre accessible à tous,

La grande différence entre ce qui a été voté en commission des affaires économiques et ce que je vous propose par cet amendement, c'est que le médiateur, s'il constate que les parties ne sont pas en capacité de se mettre d'accord,

et dénature le rôle du médiateur. En conservant la possibilité de saisir le juge des référés, ce nouvel article 3 a pour effet de bouleverser les équilibres qui ont été initialement trouvés et il nuit à la cohérence du texte. telle judiciarisation des conflits se fera nécessairement à la défaveur de la partie la plus faible, c'est-à-dire les petits producteurs, qui ne disposent pas nécessairement des moyens techniques et économiques de faire pleinement valoir leurs droits en justice. De plus, la mise en place d'un tel comité, au fait des pratiques du monde agricole, a pour objectif d'accélérer le règlement des différends pourra prendre rapidement des mesures conservatoires ou prononcer des astreintes, en cohérence avec les contraintes vécues par le secteur. Enfin, le texte issu de la commission confère au médiateur un rôle d'arbitre. Toutefois, il s'agit bien de deux fonctions distinctes, avec des missions différentes. Un tel mélange d'attributions nuit à la lisibilité du droit, mais aussi à la neutralité du règlement des litiges. Quel est l'avis de la commission ?

visent à renforcer la médiation des relations commerciales agricoles. Ils réintègrent en outre au sein du comité un représentant de la grande distribution - alors que ce comité n'examinera qu'à la marge les contrats qui concernent la grande distribution, sa cible étant le contrat entre le producteur et le premier transformateur.

témoignent de la qualité du travail de cet organisme de médiation. Nous avons donc souhaité renforcer ses pouvoirs, dans un contexte nouveau qui est celui de la contractualisation,

aller au-delà de la réflexion sur la question de la réglementation des litiges, mais en valorisant le travail du médiateur qui, une fois encore, est plébiscité par le terrain.

qui dure ... Vous dites, madame la rapporteure, que le pouvoir d'arbitre de la médiation ne sera possible que si les deux parties se mettent d'accord. Mais je vous mets mon billet que jamais les deux parties ne se mettront d'accord pour donner un pouvoir d'arbitre.

n'est pas neutre, monsieur le ministre. Je partage votre avis sur la différence entre le rôle du médiateur et celui qui consiste à rendre un avis sur l'accord qui n'a pas été trouvé.

la grande distribution restant toujours l'élément le plus fort, elle aura toujours la possibilité de sortir quand elle risque d'être condamnée ou quand elle est en tort, pour éviter d'aller jusqu'à une éventuelle pénalité. Le problème est

si un acheteur se retire d'une négociation, il n'a pas le produit, mais il ira le chercher ailleurs ; pour le producteur, s'il n'arrive pas à vendre son produit, celui-ci lui reste sur les bras, et cela devient catastrophique. Mon amendement tend, dans un premier temps, à supprimer

et l'exécution des contrats amont. Nous soutenons ce nouveau dispositif, mais nous souhaitons en préciser la composition afin que l'ensemble des parties prenantes puissent être représentées. Actuellement, le CRDCA comprend un représentant des juridictions administratives ou judiciaires, des représentants du monde agricole, que ce soit de la production ou de la transformation, et cinq membres suppléants. Nous souhaiterions que ce CRDCA soit renforcé par deux personnes. D'abord, le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM). Il nous semblerait en effet utile que cet observatoire, dont le rôle et les connaissances sont précieux, soit représenté. Puis, une personnalité représentant les associations nationales de consommateurs. C'est l'objet du présent amendement.

si les acheteurs des produits agricoles ne la justifient pas au regard des indicateurs que leur famille a validés en interprofession. En effet, il pourrait s'agir, comme le démontrent certains exemples, d'une qualification de publicité mensongère. Pour cela, il est proposé de donner au CRDCA la possibilité, sur saisine d'un opérateur ou d'une organisation professionnelle, de vérifier et valider la vérité des allégations. Il l'autoriserait, le cas échéant, à saisir la DGCCRF, pour décider des suites ou sanctions à donner.

que le médiateur se consacre exclusivement à sa fonction de médiation, dans l'intérêt des parties concernées.

Le système tel qu'il existe aujourd'hui fonctionne plutôt mal, et la rédaction actuelle pourrait encore un peu dégrader les choses. Cet amendement vise donc à envoyer un signal de fermeté dans la gestion des litiges.

Il s'agit, pour le médiateur, d'être nommé arbitre sur l'initiative des parties et non pas automatiquement. La commission a ainsi voulu donner la priorité à la volonté de résorption amiable

afin de lutter plus efficacement contre la recrudescence des allégations visant clairement à tromper le consommateur sur l'origine des produits alimentaires et, par conséquent, à les induire en erreur sur la qualité environnementale et les impacts climatiques de leur consommation alimentaire. En effet, comme cela a été souligné en commission, la consommation de produits alimentaires français est plutôt plébiscitée par les ménages et nous assistons à une multiplication des stratégies marketing de certains industriels de l'agroalimentaire qui, de manière abusive,

pourtant été supprimé en commission, au motif qu'il était satisfait par le droit en vigueur et qu'il risquait d'être contraire au droit européen. La lutte contre les allégations trompeuses sur l'origine d'un produit participe pourtant de la protection de nos agriculteurs.

Cet amendement vise à rétablir l'esprit de l'article 3 , dont la teneur a été supprimée en commission, afin de réaffirmer la nécessité de s'opposer aux pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires et d'assurer aux consommateurs une information claire et fiable. il renvoie à un décret le soin de déterminer la liste des ingrédients qui n'entreront pas dans le champ d'application de cette mesure, au motif qu'ils ne peuvent pas être produits sur le territoire français. pensent notamment au cacao, mais de nombreux exemples existent. L'article 3 , qui va dans le sens d'un renforcement de nos productions françaises et de la transparence vis-à-vis du consommateur, ne doit pas en effet être perçu comme punitif pour des filières de bonne foi qui utilisent des ingrédients et un savoir-faire français, mais qui ne peuvent tout simplement

trompeuses, tout en exemptant par voie réglementaire les produits et ingrédients primaires pour lesquels la production en France ne peut être assurée. Cette liste comprendra également des dérogations pour les cas qui conduiraient à des ruptures d'approvisionnement exceptionnelles et qui provoqueraient donc des pénuries- j'entends par là des catastrophes naturelles, des intempéries ou encore des pandémies. Prendre en considération la spécificité de certains produits et de certaines filières, ou encore l'impossibilité de se fournir dans une situation particulière, permet de trouver un équilibre entre les agriculteurs et les acteurs de l'agroalimentaire. de l'agroalimentaire. Nous devons associer toutes les parties prenantes. Les fabricants et les industriels ne peuvent être mis de côté ni entravés trop durement. N'oublions pas que l'objectif principal est d'assurer un affichage clair

Les amendements n 41 et 122 rectifié prévoient par ailleurs un décret pour tenir compte de produits comme le cacao ou le café, qui ne peuvent pas être trouvés en France. La commission, nous l'avons déjà dit, partage l'idée selon laquelle il faut renforcer l'information du consommateur face à la profusion de logos qui jouent sur l'ambiguïté du droit pour laisser penser que le produit est entièrement composé d'ingrédients d'origine française. La difficulté, mes chers collègues, c'est que vos amendements, malgré la subtilité de leur rédaction, sont toujours incompatibles avec le droit européen, qui est d'application maximale. Ils le durcissent et pourraient donc être préjudiciables à des entreprises françaises, alors même qu'une solution efficace, applicable et inattaquable est proposée par la commission à l'article 4.

» les propositions de la commission. L'un d'entre eux apporte notamment des éléments de réponse aux inquiétudes des fabricants de produits dont l'ingrédient primaire n'existe pas en France.

amendement vise donc à réintroduire le dispositif permettant de sanctionner l'utilisation du drapeau français pour des produits qui

à ce propos un mauvais souvenir, qui n'est pas si vieux : à la suite de l'initiative d'une entreprise, ce droit d'expérimentation nous a été retiré, monsieur le ministre.

ils demandent de la transparence et une meilleure rémunération pour les agriculteurs français. Renforcer l'étiquetage sur l'origine est une demande sociétale forte un affichage clair, sans équivoque, de l'origine des produits et de celle de leurs ingrédients lorsqu'il s'agit de produits transformés. Trop souvent, les étiquetages laissent penser qu'un produit est composé de matières premières agricoles françaises alors que c'est seulement l'acte de transformation- et encore -qui a lieu en France. Il convient donc d'encadrer plus strictement ces pratiques. L'apposition du drapeau français

en tenant compte des éléments apportés par la commission. Il conserve donc la publication d'un rapport sur les contrôles des pratiques commerciales trompeuses, et prend en compte les potentielles difficultés de mise en oeuvre de l'article de l'article pour des produits transformés en France à partir d'ingrédients comme le cacao, le thé ou le café. La commission des affaires économiques a souhaité remplacer l'article 3 par une demande de rapport au Gouvernement sur les contrôles réalisés par la DGCCRF sur les pratiques commerciales trompeuses liées à l'origine. Ce rapport présente un évident intérêt et l'amendement conserve aussi cette disposition. Toutefois, cela nous semble largement insuffisant. Supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, qui sanctionne le fait de faire figurer un symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients « primaires » ne sont pas français va à l'encontre de l'intérêt des agriculteurs, des consommateurs et des transformateurs qui s'approvisionnent localement. Pour prendre en compte les ingrédients exotiques, l'amendement prévoit qu'un décret précisera les produits qui pourraient exceptionnellement déroger à cette mesure, comme le chocolat ou le café. Toutefois, à la différence de l'amendement précédent, fabricants de ces produits, pour faire figurer le symbole de l'origine France, seraient tenus d'apposer de façon tout aussi visible des informations claires sur l'origine des ingrédients primaires, afin d'être totalement transparents vis-à-vis du consommateur.

l'ajout d'un décret tel que visé par le présent amendement permettra de sécuriser le dispositif par la notification obligatoire auprès de la Commission européenne. Il nous faut donc aller plus loin, malgré les difficultés d'articulation avec l'Union européenne, afin de protéger à la fois nos consommateurs, nos producteurs

partageant le souci des auteurs de la proposition de loi visant à écarter les affichages trompeurs, je considère qu'il convient néanmoins d'apporter une réponse aux PME agroalimentaires qui souhaitent légitimement valoriser la transformation réalisée en France, notamment sur des produits dont l'ingrédient primaire ne peut pas être d'origine française. C'est le

Par exemple, vous l'avez dit, monsieur le ministre, certaines marques fabriquent du café et torréfient sur notre territoire des grains importés en utilisant des méthodes de haute précision technologique donnant une qualité unique et spécifique à leurs produits. Les entreprises recourent également à des personnels qualifiés, en l'occurrence à des maîtres torréfacteurs. La nécessité d'informer les consommateurs doit conduire à une réflexion sur le flou qui existe autour des mentions « fabriqué en France » ou « origine France ». Cet amendement vise ainsi à promouvoir une valorisation de ces produits qui feraient appel à un savoir-faire français spécifique, que le consommateur est en droit de reconnaître.

Les apiculteurs français tiennent légitimement à valoriser leur production. Cela se comprend, car ils sont concurrencés par des producteurs de miels d'importation, dont beaucoup sont de mauvaise qualité. Certains de ces miels peuvent se retrouver dans des mélanges, alors même qu'il existe du miel frelaté en provenance d'Asie du Sud-Est, coupé au sucre. Les consommateurs français doivent savoir clairement ce qu'ils consomment et pourquoi certains produits sont à très bas coût. Aussi, il est urgent d'utiliser un nouveau véhicule législatif et de permettre à l'État français de publier les décrets qui mettront en oeuvre l'obligation d'étiquetage de l'origine du miel et de la gelée royale dans les mélanges.

Le présent amendement tend à corriger cet état de fait et à rendre applicables les dispositions des articles 2, 8 et 9. L'article 2 rend obligatoire l'indication du pays d'origine pour les produits composés de cacao et prévoit l'affichage, pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, de tous les pays d'origine de la récolte, indiqués par ordre pondéral décroissant sur l'étiquette. L'article 8 prévoit que les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons indiquent de manière lisible sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

car elle a été promulguée avant la fin du délai de notification à la Commission européenne, laquelle a donc refusé de se pencher sur le sujet. Aussi, plusieurs dispositions de la loi sont aujourd'hui des coquilles vides.

miel, l'amendement n° 82 rectifié ne précise pas que l'affichage doit se faire selon un ordre pondéral croissant. Or ce point a fait l'objet de nombreux débats dans cette assemblée et est attendu par l'écrasante majorité des acteurs de la filière.

notre amendement tend à revenir au principe d'un étiquetage de l'origine des ingrédients des produits transformés qui soit transparent pour le consommateur et protecteur pour le producteur.

au terme d'une consultation publique associant notamment les consommateurs et leurs représentants. En effet, la question de la rémunération de nos agriculteurs est une préoccupation partagée par tous, au-delà des acteurs de la chaîne agroalimentaire

de notre collègue Olivier Cigolotti, vise à lever les difficultés d'application des nouvelles dispositions du code de commerce aux négociations commerciales à venir. Il reporte ainsi la date d'entrée en vigueur de l'article 2, afin que les dispositions prévues par cet article puissent être applicables à un cycle complet

Les résultats des négociations de 2021 sont sans appel : alors que la rémunération des agriculteurs est restée particulièrement basse, force est de constater que les gains de productivité de l'agriculture ont été captés par d'autres, en particulier par la grande distribution. Cette loi de 2018 n'a donc pas permis de structurer le marché ; nous ne sommes guère étonnés ! La nouvelle proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans ce continuum législatif qui peine à atteindre sa cible. Je pense sincèrement que nous aurions pu aller plus loin, car, vous le savez, la situation des agriculteurs ne s'est guère améliorée- au contraire, elle a été très fragilisée par la crise sanitaire et économique que nous traversons. À l'heure où le renouvellement des générations est incertain en agriculture, comment convaincre des jeunes de se lancer dans ces métiers, dont nous avons tant besoin, s'ils n'en vivent pas correctement ? ? Comment prétendre que la transition nécessaire de notre agriculture, transition que nous souhaitons tous, est envisageable sans une juste rémunération ? Comment allons-nous permettre à nos producteurs de réaliser ces investissements ? Le texte proposé par notre collègue député était donc un rendez-vous attendu. Mais, à l'issue des débats, nous restons tous sur notre faim ! Oui, certaines mesures sont intéressantes et vont dans le bon sens, comme le meilleur encadrement des produits vendus sous marque de de distributeur, la création d'un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ou encore la sortie du prix des matières premières agricoles du cadre de la négociation tarifaire entre les industriels et les distributeurs. Mais ces avancées, nous le percevons déjà, seront insuffisantes. J'avais pourtant proposé, avec mes collègues, que des mesures concrètes soient prises pour répondre à l'écueil principal de cette proposition de loi tant que la couverture des coûts de production des agriculteurs ne sera pas garantie dans les négociations commerciales, leur revenu ne pourra pas l'être non plus.

Je pense à la régulation des marques de distributeur, au rétablissement sous condition de l'article 3 , visant à défendre le, aux dispositions relatives à l'information sur l'origine des viandes. Nous regrettons toutefois un certain nombre de reculs, tout particulièrement la réécriture de l'article 2, qui a affaibli la transparence de nos produits.

ce que n'a pas permis la loi Égalim 1 -en sécurisant la part agricole dans les tarifs du fournisseur, pour « construire le prix en marche avant » dans le cadre d'une contractualisation obligatoire

L'industriel n'est rien sans l'agriculteur, mais la grande distribution n'est rien sans l'industriel. À la fin des fins, le consommateur a aussi besoin des circuits de distribution. Comme je le disais hier dans mon propos introductif, c'est toute la chaîne